La séance est reprise. Nous reprenons l'examen de la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

de la 5G. Le rapport du Haut Conseil pour le climat a indiqué que la 5G pouvait induire des émissions de gaz à effet de serre, qui doivent être anticipées et maîtrisées. précisé que ces émissions dépendraient de plusieurs facteurs : modalités de déploiement retenues par les opérateurs, renouvellement des terminaux de 5G ou encore évolution de l'offre de services numériques et de leurs usages potentiels.

pour poser les fondements d'une nouvelle approche, avec davantage de transparence et une plus grande association de la représentation nationale. Il nous semble crucial de réconcilier élus et citoyens avec cette nouvelle technologie et de relancer sereinement le débat public sur son déploiement.

au travers de cet amendement, que le rapport détaille les mesures proposées pour informer, sensibiliser et responsabiliser les usagers- particuliers et entreprises -aux bonnes pratiques permettant de réduire l'empreinte environnementale du numérique.

Je ne voudrais donc pas que l'on se retrouve dans une situation comparable avec la 5G, avec des enjeux encore plus importants, notamment en matière de compétitivité industrielle de notre pays.

: La parole est à M. Jacques Fernique. Cet amendement d'appel vise à demander au Gouvernement d'intégrer des objectifs propres au numérique dans la fameuse stratégie nationale bas-carbone Cette stratégie définit un « budget carbone », qui correspond à des plafonds d'émission de gaz à effet de serre, que différents secteurs ne doivent pas dépasser. Elle a donc un rôle structurant dans les politiques publiques mises en place pour atteindre nos objectifs environnementaux. Compte tenu de l'impact carbone grandissant du numérique, il paraît essentiel que ce dernier soit pris en compte dans les orientations de la France et dans les objectifs visant à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le numérique ne saurait être tenu hors du champ de la SNBC,

C'est une piste que nous jugeons intéressante ; nous avons eu l'occasion de l'étudier. Néanmoins, l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, qui définit la stratégie nationale bas-carbone,

en son article 4, aux seuls usages numériques des entreprises, ce qui exclut les biens exploités ou commercialisés. Le présent amendement vise donc à inclure, au sein des déclarations de performance extrafinancière des grandes entreprises, outre l'évaluation de l'impact environnemental des biens et services numériques utilisés en interne, ceux qui sont exploités ou commercialisés.

à la position de la commission. Quel est l'avis de la commission ? Le fait de prévoir une évaluation de l'impact environnemental des biens et services numériques dans le bilan RSE entre bien dans le champ de la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui doit communiquer ces informations, dans le cadre de son rapport de gestion.

Il complète donc opportunément l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; il s'agit à nos yeux d'une évolution extrêmement positive même si elle ne touche pas toutes les entreprises.

travers notamment de la création d'un crédit d'impôt en faveur de la numérisation durable ; il s'agit d'accompagner ces entreprises dans la mise en place d'une stratégie de transformation numérique incluant l'objectif de sobriété numérique.

La méthode actuelle du bilan carbone ne comprend pas le bilan lié aux activités numériques. Tel est l'objet de notre amendement. Quel

en faire une obligation pour tous ces acteurs peut paraître un peu trop lourd. Il serait peut-être plus efficace d'intégrer cet enjeu de manière plus lisible dans le cadre de la méthodologie d'élaboration de ces bilans, afin que ces derniers puissent aborder ce point de manière systématique. Cela rejoindrait d'ailleurs les travaux en cours visant à définir une méthodologie d'évaluation de cette empreinte. Nous nous positionnons plus dans une logique d'accompagnement que dans une logique contraignante. La commission a donc émis un avis défavorable

L'article 5 du texte instaure un crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises destiné à prendre en charge 50 % des dépenses d'accompagnement pour la mise en place d'une stratégie de transformation numérique numérique incluant la sobriété numérique, mais aussi les dépenses d'acquisition d'équipements numériques reconditionnés. Afin d'encourager la gestion des ressources informatiques et des matières premières nécessaires à la fabrication des biens, le présent amendement tend donc à rendre éligibles à ce crédit d'impôt les dépenses destinées au recours à des équipements numériques issus de l'économie de la fonctionnalité.

à la réalisation d'études d'impact environnemental des services numériques, les frais d'accompagnement pour la mise en place d'une stratégie de transformation numérique de l'entreprise et les dépenses destinées à l'acquisition d'équipements numériques reconditionnés. Cet amendement vise à élargir les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt aux dépenses destinées au recours à des équipements numériques issus de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité peut se définir comme un système économique

La limitation du renouvellement des terminaux, dont la fabrication et la distribution représentent, je le rappelle, près de 70 % de l'empreinte carbone du numérique en France, constitue un jeu écologique majeur. en 2018 par une enquête pour obsolescence programmée et tromperie, le fabricant Apple a reconnu qu'il altérait volontairement les performances de ses iPhone à batterie

il permet de rendre opérant le délit d'obsolescence programmée, aujourd'hui complètement inapplicable, en supprimant l'un des deux critères requis pour le caractériser. En effet, à ce jour, l'article L. 441-2 du code de la consommation définit l'obsolescence programmée par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement prévoit la suppression d'un des deux critères d'intentionnalité, celui de l'intention délibérée d'augmenter le taux de remplacement du terminal, afin que l'obsolescence programmée soit définie, plus simplement, comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie ». Force est de constater que le standard de preuve actuellement requis pour caractériser la pratique d'obsolescence programmée se révèle souvent trop élevé et peu opérant, comme l'a illustré le dossier Apple. Dans sa réponse au questionnaire adressé par les rapporteurs, la DGCCRF indique en effet que les dossiers qu'elle a instruits n'ont pu être menés à bien sur ce fondement juridique, faute de réunir les éléments suffisants permettant de caractériser le délit. Je veux donc saluer les travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ayant abouti

afin de permettre à l'utilisateur d'installer seulement celles qui n'entraveront pas le fonctionnement de son bien, rendant celui-ci prématurément obsolète. Si la conformité d'un bien est définie à l'article L. 217-5 du code de la consommation, il convient de lever toute ambiguïté et de sécuriser l'application de cet article. amendement précise que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l'exclusion des mises à jour évolutives. Cette distinction est celle qui est retenue par la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 « Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs ». Quel est

pour signaler que, du point de vue du Gouvernement, les articles 8 et 9 sont déjà satisfaits, notamment dans le cadre de la transposition en cours des directives 2019/770 et 2019/771 de l'Union

qui, aujourd'hui, représenteraient déjà près de 10 % du marché. La présente proposition de loi prévoit de diminuer le taux de TVA appliqué à ces produits, ce qui est une très bonne chose.

totalement l'objet de cet amendement : si nous voulons développer cette filière essentielle, il faut lever un certain nombre de freins, au premier rang desquels la confiance en la fiabilité et en la qualité du produit reconditionné. C'est pourquoi il convient de prévoir des garanties de traçabilité de ces produits, afin que le consommateur puisse avoir la garantie qu'un certain nombre de prescriptions liées à la qualité du produit ont été respectées, ainsi que des informations sur la provenance et le lieu de reconditionnement de ces produits. L'avis de la commission est donc favorable. Quel est l'avis du Gouvernement du Gouvernement ? Le présent amendement tend à compléter l'article L. 122-21-1 du code de la consommation, qui prévoit que les conditions d'utilisation de la mention « reconditionné » ou « produit reconditionné » sont précisées par décret. du présent amendement apporterait de nouvelles exigences pour les produits électriques et électroniques, pour l'utilisation de ces mentions en matière de conformité, de contrôle du fonctionnement, de suppression des données, d'affichage des pays de provenance et de reconditionnement du produit. Or l'article en question concerne tous les produits reconditionnés, et pas seulement ces deux catégories d'équipements. Ces éléments font, d'ores et déjà, l'objet d'un projet de décret en cours d'élaboration par le Gouvernement. Il ne nous semble donc pas nécessaire de modifier la loi. Par conséquent, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

nous proposons ainsi de renforcer cet aspect, en faisant de la garantie légale de conformité un outil au service de l'allongement de la durée de vie des produits. La garantie légale est le premier levier à la disposition du consommateur pour se protéger des pannes et de l'obsolescence accélérée. Pour que cet outil contribue à la transition vers une économie circulaire, il doit favoriser la réparation au remplacement des biens. Au travers de cet amendement, nous proposons ainsi plusieurs dispositions

est l'avis de la commission ? Cet amendement tend, par des moyens très hétérogènes, à ce que la réparation soit privilégiée par rapport au remplacement dans le cadre de la garantie légale de conformité. Premièrement, la partie de l'amendement visant à ce que la réparation soit rendue prioritaire par rapport au remplacement est en partie satisfaite par les modifications introduites par la loi AGEC. Cette dernière prévoit en effet que, à compter de 2022, dès lors que le consommateur fera le choix de la réparation, mais que celle-ci ne sera pas mise en oeuvre par le vendeur, le consommateur pourra demander le remplacement du bien, qui s'accompagnera, dans ce cas, d'un renouvellement intégral de la garantie légale de conformité. Le vendeur est donc fortement incité à privilégier la réparation. Deuxièmement, l'obligation de justification par écrit au client du fait que la réparation entraînerait un coût disproportionné introduirait une contrainte pour le vendeur, sans, pour autant, que le droit du consommateur soit réellement accru. Troisièmement, l'obligation de remise d'un rapport au client avec le détail des réparations effectuées et la nature des pièces détachées installées ne nous semble pas relever du cadre juridique relatif à la garantie légale de conformité.

sur les réparations. Nous avions déjà proposé, lors de l'examen de la loi sur l'économie circulaire, la mise en oeuvre d'une garantie générale de bon fonctionnement de six mois sur les biens réparés en dehors de la garantie légale, c'est-à-dire la catégorie « A+ ». Il s'agit ainsi d'aller au-delà de ce qui est actuellement prévu par la loi, c'est-à-dire, en cas de réparation dans le cadre de la garantie de conformité, une extension de celle-ci de six mois et la réinitialisation de la garantie en cas de remplacement. Nous estimons que le législateur peut aller encore plus loin. En effet, dans 60 % des cas de pannes, le consommateur n'essaye pas de faire réparer son produit. Pourtant, dans une économie circulaire, la réparation et le reconditionnement doivent être encouragés : ces solutions permettent d'allonger la durée de vie des produits tout en étant vertueuses sur le plan environnemental. Actuellement, une fois la garantie d'un bien dépassée, l'usager peut faire le choix de se tourner vers un réparateur professionnel. Toutefois, à la suite d'une réparation, une défaillance peut survenir sans aucune protection juridique pour le client, ce qui peut le dissuader d'avoir recours à cette solution. Nombre de réparateurs indépendants offrent déjà une garantie de six mois à leurs clients. Afin de généraliser cette pratique, de protéger les consommateurs et de les inciter à réparer leur produit plutôt qu'à en racheter un neuf, une garantie légale sur les actes de réparation professionnelle doit pouvoir être offerte pendant au moins six mois par tous les réparateurs. Quel

programmée du produit. Il s'agit de deux informations complémentaires nécessaires à la bonne information du consommateur, lui permettant de faire des choix éclairés et de favoriser l'achat de biens durables et réparables.

Par souci de clarté, il ne nous semble pas pertinent de multiplier les sources d'information pour le consommateur. Par ailleurs, je note que la rédaction de cet amendement conduirait à imposer cette obligation à l'ensemble des équipements électriques et électroniques, et pas seulement aux équipements numériques, seuls concernés par cette proposition de loi. La commission demande donc le retrait de cet amendement

un réel compteur d'usage sur certains produits, notamment sur les équipements électroniques et numériques. Aujourd'hui, les compteurs d'usage ne sont pas obligatoires. Nous considérons que ce serait un plus, une garantie,

au niveau du marché unique. Nous ne sommes donc pas favorables à un dispositif national. Notons, cependant, que dans une résolution du 25 novembre 2020 le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la mise en place de compteurs d'usage à l'échelle européenne. Il serait donc intéressant de porter ce sujet à ce

Cette proposition vise, en effet, la fixation d'objectifs spécifiques de recyclage, de réemploi et de réparation pour certaines catégories d'équipements numériques. Elle est articulée avec les avancées opérées par la loi AGEC et relatives au fonds de réemploi et de réutilisation, ainsi qu'au fonds de réparation. Je tiens à annoncer à la Haute Assemblée que ces mesures seront intégrées dans les cahiers des charges des éco-organismes de il nous semble essentiel de laisser au dispositif le temps de se mettre en place et d'analyser son efficacité avant de modifier ses règles. C'est pourquoi nous sommes défavorables à l'article et, partant, à cet amendement rédactionnel.

de réemploi et de réparation pour certaines catégories d'équipements numériques, objectifs fixés par le cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques. Or l'entrée en vigueur de tels objectifs a été décalée par la commission en 2028, soit dans sept ans. Pour justifier ce report, cet article s'appuie sur les nombreuses évolutions législatives apportées par la loi relative à l'économie circulaire. Certes, de nouvelles obligations sont imposées, notamment la création d'un fonds de réemploi ainsi que des objectifs plus ambitieux de réemploi dans le cahier des charges

Reporter de six ans l'obligation définie serait un très mauvais signal envoyé dans la lutte contre les déchets liés aux équipements électroniques et numériques. Nous proposons donc une entrée en vigueur au 1 janvier 2022. Quel l'avis de la commission ? L'article 12 prévoit, dans le prolongement de ce qui a été fait dans la loi AGEC, que les cahiers des charges des éco-organismes de la filière DEEE fixent des objectifs spécifiques de recyclage, de réemploi et de réparation pour certaines catégories d'équipements numériques. L'idée est de cibler les smartphones et tablettes, afin d'éviter qu'ils ne soient noyés dans des objectifs communs pour toute la filière.

En effet, une telle modification est loin d'être anodine et nécessiterait de mettre en oeuvre de nouveaux flux distincts, lourds à organiser. Le nouvel agrément prenant en compte toutes les modifications de la loi AGEC doit être adopté début 2022. Il serait particulièrement difficile d'imposer aux acteurs d'ajouter une nouvelle disposition. Nous ignorons, en effet, quand le texte sera définitivement adopté : seulement quelques mois ou quelques semaines avant le nouvel agrément. En outre, le processus de renégociation du nouvel agrément est long

leur recyclage ou leur réutilisation. Nous savons tous que, dans le domaine de l'économie circulaire, la réduction des déchets et le développement de la valorisation des équipements numériques apparaissent comme une priorité à étudier et à expérimenter. établir sur le fondement du volontariat à l'échelle des collectivités territoriales semble mieux adapté pour déterminer quel procédé de recyclage fonctionne le mieux. À ce titre, la consignation de certains équipements numériques, afin d'accroître le taux de collecte des équipements réemployables avant qu'ils ne perdent leur valeur d'usage et ne deviennent des déchets, serait un progrès notable dans la réduction de l'empreinte carbone. Cela allongerait la durée de vie des produits, tout en réduisant les déchets d'équipements électriques et électroniques.

En premier lieu, les collectivités pourraient, d'ores et déjà, prévoir ce type de mesures : soit en partenariat avec des entreprises ou avec l'éco-organisme en charge de la collecte de ces équipements ; soit un système de gratifications que rien ne leur interdit, à ce jour, de déployer.

Même avis, madame la présidente. Fernique. Cet amendement vise à proposer au Gouvernement d'élaborer une étude d'impact et de faisabilité, afin d'améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques, actuellement très peu recyclés. Au regard de la complexité de la mise en oeuvre de tels dispositifs, mais également de la nécessité de réduire le gaspillage et les déchets des équipements numériques, il est essentiel d'évaluer toutes les solutions envisageables pour leur réemploi. Ce rapport pourrait étudier la possibilité d'une mise en place de consignations d'équipements numériques. Il pourrait également considérer l'opportunité de passeports-produits, c'est-à-dire d'un dispositif d'identification unique de l'équipement permettant d'assurer la traçabilité et la disponibilité d'informations sur les caractéristiques des produits et de comptabiliser le flux de réemploi ou reconditionnement en parallèle du flux de recyclage. À ce titre, dans son plan d'action d'économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive, la Commission européenne, annonce la mise en place de passeports numériques. Enfin, ce rapport pourrait étudier l'installation ou l'élargissement d'un dispositif de collecte des déchets d'équipements électriques ou électroniques dans certains magasins. Une étude sur la faisabilité de mise en oeuvre de tous ces dispositifs paraît très opportune pour un recyclage efficace des équipements numériques.

numériques. La structuration d'une filière de recyclage et de terminaux numériques et les enjeux de développement du réemploi et de la réutilisation de ces biens sont essentiels pour limiter le renouvellement excessif. Une fois n'est pas coutume, nous émettons un avis favorable sur cet amendement.

est à M. Hervé Gillé. La commission a adopté un amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dont l'objectif est de faire de l'achat public un levier pour réduire l'empreinte carbone du numérique. Ainsi, le texte de la proposition de loi inscrit désormais la politique d'achat dans une démarche de durabilité des produits et de sobriété numérique dans le cadre des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Ces schémas sont actuellement applicables aux collectivités dont le montant annuel des achats dépasse le seuil de 100 millions d'euros, hors taxes. cette obligation concerne uniquement les très grandes collectivités. Selon Bercy, 160 organisations seulement seraient concernées par cette obligation, ce qui est peu. Pourtant, la forme de ce schéma est libre et peut s'appuyer sur le plan national d'action pour les achats publics durables, le PNAAPD. Une nouvelle version de ce plan est d'ailleurs annoncée pour début 2021. Comme l'a rappelé le commissariat général au développement durable, le 10 décembre dernier, l'achat public doit jouer un rôle clé et vertueux dans la relance. La commande publique doit intégrer davantage de durabilité, davantage d'enjeux sociaux et environnementaux, pour avoir un effet plus transformant. Par ailleurs, la feuille de route présentée en 2018 par le Gouvernement pour l'économie circulaire- il s'agit de -prévoit d'abaisser le seuil à partir duquel devient obligatoire le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Ainsi, notre amendement tend à concrétiser cette mesure en introduisant un seuil légal fixé à un montant total annuel des achats à 75 millions d'euros, au lieu des 100 millions d'euros actuellement fixés par Tel est le sens de notre amendement, dont l'adoption devrait inciter davantage de collectivités à s'interroger sur leur stratégie d'achat et à intégrer l'enjeu de durabilité des produits et de sobriété numérique.

les enjeux de durabilité des produits et de sobriété numérique dans les schémas de promotion des achats publics responsables. Aujourd'hui, ces schémas doivent être élaborés par les collectivités dont le montant annuel total des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire : 100 millions d'euros. La pertinence de ce seuil particulièrement élevé se pose en effet. Vous l'avez souligné, le Gouvernement avait indiqué, au moment des débats sur la loi AGEC, que la révision du plan national d'action pour des achats durables

puis de durabilité à moyen terme, pour l'acquisition de leurs produits numériques. L'indice de réparabilité est entré en vigueur depuis le 1janvier 2021. Certes, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à disposer d'un an pour s'adapter. Cependant, afin de les inciter à adopter le plus rapidement cet indice,

Nous connaissons le sort des amendements visant à instaurer des taux de TVA réduits : en effet, nous avons tenté à plusieurs reprises d'abaisser le taux de TVA des services de réparation, tout en ayant conscience des difficultés que pose actuellement l'annexe III de la directive TVA du 28 novembre 2006, qui établit une liste limitative des biens et services pouvant en bénéficier. Toutefois, la brèche est ouverte par le présent texte. En conséquence, nous proposons d'élargir le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % aux produits issus du réemploi ou de la réutilisation, ainsi qu'aux services de mise à disposition de l'usage des biens moyennant facturation, c'est-à-dire des biens issus de l'économie de la fonctionnalité. une négociation doit avoir lieu dans le cadre de la révision de la directive européenne de 2006, elle doit permettre d'envoyer un signal prix positif au bénéfice de ces biens plus vertueux, qui permettront de limiter l'impact environnemental du numérique.

une TVA réduite pour l'acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés et pour les services de réparation de biens comportant des éléments numériques. La mission d'information dont ce texte est issu avait en effet considéré que de tels taux de TVA réduits pourraient contribuer à renforcer l'attractivité des offres issues du reconditionnement et de la réparation et, ainsi, à limiter le renouvellement des terminaux. De tels taux concourraient également à la structuration dans les territoires d'un écosystème industriel du reconditionnement et de la réparation. Néanmoins- M. Gold l'a lui-même souligné -, nous sommes conscients que, en l'état actuel du droit européen une telle modification se heurte à l'impossibilité pour les États membres de fixer un taux réduit pour des biens et des services qui ne figurent pas dans l'annexe de la directive TVA.

nous sommes défavorables à l'article 14 et, par extension, à l'amendement

des produits reconditionnés, dont les smartphones et ordinateurs, ayant déjà fait l'objet d'une première mise sur le marché en Europe. En effet, la rémunération pour copie privée est acquittée sur les produits neufs lors de leur mise en circulation en Europe. Or un produit ne peut faire l'objet que d'une seule mise en circulation au sens de l'article 1245-4 du code civil. Ainsi, cette rémunération ne saurait s'appliquer aux produits reconditionnés qui proviennent d'Europe, puisque la redevance ne doit être payée qu'une seule fois sur un même produit. En outre, l'application de cette obligation aux produits reconditionnés ferait peser une menace sur un secteur en développement, qui apporte une contribution majeure à l'essor d'une économie numérique plus circulaire et plus vertueuse. Enfin, si ces produits numériques reconditionnés devaient être soumis à une telle redevance, le coût supplémentaire serait supporté par les consommateurs eux-mêmes. En conséquence, l'achat de produits neufs à faible coût, mais de moindre qualité technique et présentant un plus fort impact environnemental, pourrait être favorisé aux dépens de produits reconditionnés en Europe.

d'une perte de recettes hypothétique. Cela étant, la question se pose et elle va sans doute faire débat : est-il pertinent que les biens reconditionnés contribuent au financement d'activités culturelles ?

Autrement dit, cet assujettissement annulerait presque intégralement la baisse des taux de TVA sur les biens reconditionnés, que nous avons souhaité introduire à l'article 14. De plus, ces dispositions n'empêcheraient pas le prélèvement

la compétitivité des activités de reconditionnement nationales et européennes aux dépens du reconditionnement extraeuropéen. Je le répète, selon les

Face à ces pratiques, la Convention citoyenne pour le climat a, elle aussi, formulé des propositions pour une consommation plus sobre et plus vertueuse sur le plan environnemental. L'un des leviers d'action serait la régulation de la publicité : il s'agirait de réduire les incitations à la surconsommation. D'ailleurs, depuis le 1 janvier 2021, toute publicité visant à promouvoir la mise au rebut

encourageant le renouvellement des terminaux, notamment des smartphones. Nous proposons de compléter ce dispositif pour améliorer la transparence de l'information fournie aux utilisateurs

accès à internet doit être assortie d'un message de sensibilisation faisant la promotion d'un numérique responsable. La liste, l'énoncé et les modalités de diffusion de ces messages valorisant les bonnes pratiques d'usage

la logique suivie est différente. Le simple fait d'acheter un téléphone portable ou de souscrire un abonnement pour un forfait mobile ne doit pas être perçu, en soi, comme de nature à aggraver la pollution numérique.

premières rares. Ainsi, nous estimons qu'il convient d'aller vers une standardisation des chargeurs d'appareils électroniques pour éviter leur remplacement systématique. D'ailleurs, l'Europe s'engage dans cette voie.

En 2009, la Commission européenne s'emparait déjà du sujet et, deux ans plus tard, elle arrivait à réduire à trois le nombre de types de chargeurs disponibles sur le marché : le micro USB, l'USB-C et le lightning,

malgré des progrès considérables et rapides réalisés par le secteur. C'est la raison pour laquelle la proposition de loi offre la possibilité de supprimer les forfaits mobiles comprenant un accès illimité données. Or l'effet de cet article sur l'empreinte environnementale du numérique sera marginal, alors qu'il sera bien réel pour les ménages précaires et pour nos concitoyens qui ne disposent pas d'une connexion fixe wifi cette mesure sera indolore pour les ménages les plus aisés, ce qui réduira son efficacité. Alors que la couverture en très haut débit s'améliore progressivement, que nos concitoyens accèdent enfin à la 4G dans certains territoires, on leur ferait payer plus chèrement leur forfait.

président de l'Arcep : « La nécessaire sobriété du numérique ne doit pas s'entendre comme la limitation des échanges en ligne. La crise a montré combien ces échanges étaient cruciaux à la vie de la Nation, et nulle autorité ne pourrait s'ériger en juge des bons ou des mauvais usages dans la démocratie. La profusion d'internet doit rester une source inépuisable de vitalité, d'expression et d'innovation ». Il ne s'agit donc pas de ne rien faire face à l'augmentation de la demande en consommation de données, mais nous préférons privilégier la pédagogie à la contrainte et à l'application d'une disposition pénalisante pour l'ensemble des utilisateurs, sans égard pour le contexte de l'utilisation des réseaux mobiles.

à privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. Il est articulé, à ce titre, à l'article 13 de la loi

Pourquoi avions-nous choisi d'aller dans cette direction ? Nous avions constaté que les réseaux mobiles sont beaucoup plus énergivores que les réseaux fixes : le simple visionnage d'une vidéo en 4G est quatre fois plus consommateur qu'un visionnage en wifi Je rappelle également que la consommation des réseaux mobiles est en grande partie proportionnelle aux usages qui en sont faits, ce qui n'est pas le cas des réseaux fixes. Ces réalités sont souvent méconnues des Français, qu'elles expliquent en grande partie l'explosion du trafic de données mobiles- + 30 % par an -, qui jouera un rôle important dans l'accroissement considérable des impacts environnementaux des réseaux mis en avant dans notre rapport d'information. Je rappelle ainsi que la consommation énergétique des réseaux pourrait croître de 75 % d'ici à 2040. Des forfaits mobiles dont la tarification serait totalement décorrélée des données mobiles consommées ne nous semblent donc pas souhaitables, car ils annulent le message qui pourrait être adressé au consommateur visant à privilégier une connexion wifi à une connexion mobile. Nous notons également que ces forfaits constituent un biais tarifaire en faveur des plus gros consommateurs aux dépens des plus petits, qui correspondent souvent aux catégories de revenus les plus modestes. On sait, en effet, que ces personnes n'ont souvent pas les moyens de souscrire à des forfaits proposant des plafonds élevés de données ou à des forfaits illimités. Forts de ce constat, nous avons finalement préféré, dans le cadre de cette proposition de loi, laisser les opérateurs trouver les modalités, notamment tarifaires, susceptibles d'inciter les consommateurs à privilégier une connexion wifi. Les engagements contraignants que les opérateurs devront prendre sur le fondement de l'article 23 pourront notamment inclure une tarification des forfaits mobiles plus incitative.

de demander aux utilisateurs de faire en sorte d'utiliser les réseaux fixes, donc la wifi, plus que les réseaux 4G,

Pourtant, dans les zones rurales en particulier, il arrive que cette connexion soit insuffisante, voire endommagée, sur le réseau filaire cuivre, malgré les engagements des opérateurs à réparer les lignes défectueuses. Le présent amendement a donc pour objet de garantir la possibilité pour tous les consommateurs de se tourner vers un réseau filaire ou cuivre en bon état de fonctionnement. Quel

Comme le notent très justement les auteurs de cet amendement, la dégradation du réseau fixe pousse bien souvent nos compatriotes à se connecter au réseau mobile, beaucoup plus consommateur d'énergie, pour avoir accès à internet. En la matière, un cadre de régulation existe déjà : en tant qu'opérateur historique, Orange a été chargé de fournir le raccordement et le service sur ce réseau par un arrêté ministériel de novembre 2017. Sur ce fondement, l'Arcep avait mis en demeure d'améliorer sa qualité de service sur le réseau cuivre, après avoir constaté une importante dégradation. L'Arcep a, depuis lors, salué les efforts d'Orange pour l'amélioration du service universel.

on ne peut pas leur dire d'attendre la fibre pendant encore des années. Je profite de cet amendement pour vous demander de nous aider. On ne peut pas laisser des gens sans un accès filaire cuivre. Or c'est un service de base que l'on ne fournit pas à tout le monde sur le territoire. Ce n'est pas acceptable en France ! Je mets

à M. Hervé Maurey. J'ai présenté tout à l'heure des amendements qui visaient à limiter le renouvellement des terminaux. J'en viens maintenant à des amendements tendant à inciter à des pratiques plus vertueuses en matière environnementale. C'est le cas de cet amendement n° 54 rectifié. L'article 16

qui vise à rendre obligatoire l'écoconception des sites pour l'ensemble des fournisseurs de contenus, soit pour l'ensemble des personnes publiques et privées diffusant des contenus sur internet. En ce qui concerne l'amendement n° 54 rectifié, l'article 16 prévoit qu'un référentiel de l'écoconception soit respecté par les plus grands fournisseurs de contenus. Nous estimons que ce référentiel pourra parallèlement servir de référence aux acteurs qui ne sont pas assujettis à cette obligation, mais qui seraient désireux de s'engager sur le chemin d'une conception numérique responsable, notamment les sites des services publics.

En effet, nous avons été informés que des travaux, associant notamment l'Ademe, étaient en cours pour élaborer un référentiel général de l'écoconception, comme le prévoit le présent article. L'avis de cette dernière serait donc bienvenu pour élaborer le décret qui devra définir les grandes lignes de ce référentiel.

et de certaines entreprises. Le report à 2023, proposé en commission des affaires économiques et introduit en commission du développement durable, n'est pas souhaitable, dans la mesure où il existe d'ores et déjà beaucoup de matière pour établir ce référentiel. Pourquoi attendre ? Il y aurait une certaine logique à se lancer immédiatement. Il est important de créer des habitudes,

qui provoquent un gaspillage de ressources naturelles et d'énergie. C'est le cas, par exemple, à Paris, dans les transports en commun et dans les gares, mais aussi dans bien d'autres métropoles de France. un panneau publicitaire numérique consomme sept fois plus qu'un panneau d'affichage classique rétroéclairé et treize fois plus s'il comporte deux faces. Un écran de deux mètres carrés consomme, par exemple, 6 800 kilowattheures par an, soit la consommation d'un couple avec un enfant. donc complètement à l'encontre des objectifs de sobriété. Le Réseau de transport électrique, RTE, dans son bilan annuel de novembre 2019, les a lui-même qualifiés de « superflus » et de « non prioritaires répond aussi à un impératif de santé publique : l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans des lignes directrices publiées en avril 2019, comme le Défenseur des droits, dans un rapport publié en 2018, ont alerté sur les effets nocifs de l'utilisation de toute forme d'écran pour les enfants de moins de six ans. Ces écrans génèrent une surcharge cognitive au quotidien et nuisent au développement intellectuel. Les études s'accumulent sur ce sujet et recommandent d'en proscrire l'usage. Mes chers collègues, la transformation de nos villes en gigantesques panneaux publicitaires numériques est un sujet majeur. Ce texte de loi sur le numérique offre aussi l'occasion de légiférer, enfin, sur cette problématique, alors qu'une majorité de Français souhaite voir disparaître

Par ailleurs, nous proposons que les publicités numériques situées dans les vitrines des magasins soient intégrées à la législation concernant l'espace public, afin de réguler leur implantation. promenez tous dans nos villes et vous savez donc que, aujourd'hui, nous sommes agressés en permanence par ces panneaux numériques, parce que notre cerveau est conditionné pour regarder tout ce qui bouge. Nous sommes donc forcément

sur les voies de circulation publique- dans les aéroports, les gares, les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Cette interdiction s'appliquerait également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsqu'elles sont visibles depuis la voie publique, mais ne s'appliquerait pas aux panneaux d'information publique non commerciale et aux panneaux indispensables à l'intérêt général. Ce sujet a déjà suscité de larges débats, notamment lors de l'examen de la proposition de loi déposée par la députée Delphine Batho le 11 février dernier à l'Assemblée nationale. D'une manière générale,

considérant qu'il ne constitue pas le vecteur approprié pour ce type de disposition. Ces amendements visent à interdire sous une forme ou sous une autre la publicité numérique dans l'espace public. Nous considérons

pouvoir en la matière. Le chapitre 2 de l'avant-projet de loi Climat comporte également des mesures visant à réguler la publicité dans le but de limiter les incitations à la consommation : il prévoit notamment des mesures de décentralisation du pouvoir de police de la publicité, qui serait ainsi exercé par le maire, que la commune dispose ou non d'un règlement local de publicité, ou encore des dispositions permettant d'encadrer davantage la publicité dans le cadre des règlements locaux de publicité, notamment à l'intérieur des vitrines. Par ailleurs, il nous semble inopportun d'intégrer à ce stade de l'examen de notre texte, c'est-à-dire sans avoir du tout étudié ce champ de la pollution numérique ni même entendu les acteurs de ce secteur,

Le CSA a exprimé le souhait d'accompagner les transformations profondes suscitées par la lutte contre le réchauffement climatique. Compte tenu de l'impact environnemental du secteur audiovisuel, notamment dans ses composantes de diffusion

Cet amendement vise à prévoir que le rapport annuel du CSA comprenne un bilan de la mise en oeuvre par les éditeurs et les distributeurs de services des mesures de nature à limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'audiovisuel au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas-carbone et conformément aux engagements internationaux de la France, et les recommandations qu'il a émises pour remédier aux manquements constatés.

la proposition de loi, nous avons pour l'instant fait le choix de confier cette régulation à l'Arcep, tout en consacrant le rôle de l'Ademe dans la production de données et de connaissances sur le sujet. Par ailleurs, nous n'avons pas consulté le CSA dans le cadre de nos travaux ; nous ne sommes donc pas

M. Gilbert-Luc Devinaz. La sensibilisation des consommateurs à l'impact environnemental de leurs usages numériques est un axe essentiel pour inciter à la sobriété des comportements. Elle passe par une information transparente sur l'impact carbone des consommations de vidéos. Notre amendement vise donc à instaurer une information du consommateur sur l'indice environnemental lié au stockage et au visionnage des vidéos. Pour plus d'efficacité, il est proposé qu'un décret fixe les caractéristiques des contenus visés par cette mesure, notamment en fonction de leur poids. Si cette prise de conscience par les consommateurs de l'impact de leurs usages numériques les plus énergivores est essentielle, elle doit s'accompagner d'une évolution des pratiques des professionnels, notamment des grandes plateformes de.

à l'instauration d'un indice d'impact environnemental, probablement lourd à mettre en oeuvre, une obligation d'information sur la quantité de gaz à effet de serre qui est associée au visionnage d'une vidéo. J'en viens

l'utilisateur quant à la quantité de gaz à effet de serre émise lors de l'utilisation de tout type de services de communication au public en ligne nous semble constituer une obligation trop générale, pesant sur un trop grand nombre d'acteurs et pour une diversité d'usages qui rendrait difficile l'établissement d'une méthodologie appropriée

que l'utilisateur soit informé des effets des vidéos visionnées sur les sites de VOD. En particulier, il nous paraît utile que soient distinguées les émissions de gaz à effet de serre associées au visionnage d'une vidéo selon le niveau d'affichage et de résolution proposé et selon le type de connexion utilisé. Par ce biais, l'utilisateur pourra par exemple prendre conscience du fait que le visionnage d'une vidéo en 4G est quatre fois plus consommateur en énergie

initiale. Quel est l'avis de la commission ? Les modifications introduites par la commission à l'article 16, visant à ce que soit créé un référentiel général de l'écoconception, vont plus loin que ce que préconisait l'article 17 dans sa version initiale au lieu de demander l'intégration dans le rapport d'informations relatives aux stratégies de captation de l'attention, l'article 16 inclut directement dans le référentiel de l'écoconception les critères qui limiteront le recours à ces stratégies.

Au sein de la commission, nous avons souhaité privilégier une régulation s'appuyant sur une obligation générale d'écoconception des services numériques et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif, créé à l'article 16, plutôt que de recourir à des interdictions législatives. les mesures législatives sont rigides et lentes d'évolution, des caractéristiques incompatibles avec la multitude des usages numériques et leur mutation constante du fait des nombreuses innovations que connaît le secteur. Il nous semble donc que les dispositions visées par les articles 18, 19 et 20 supprimés seront mieux servies par un référentiel unique, qui pourra définir des règles sur une palette de sujets bien plus large. Nous rappelons que les sujets visés dans les articles 18, 19 et 20 de la proposition de loi seront encadrés par le référentiel, puisque l'article 16 précise que les critères du référentiel devront notamment concerner « les règles relatives à l'ergonomie des services numériques, ainsi qu'à l'affichage et la lecture des contenus multimédias Nous rappelons également que, si ce référentiel n'est pas de nature législative, l'obligation d'écoconception l'est et sera vérifiée par l'Arcep, qui disposera d'un pouvoir de sanction. Il nous semble contre-productif de rétablir en parallèle de ce référentiel des interdictions législatives qui rendraient la régulation en vigueur moins adaptative à la mutation constante des pratiques numériques. J'émets donc un avis défavorable

la présidente. L'amendement n° 26 rectifié est retiré. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance pour achever l'examen

M. Cédric Perrin. Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent que les centres de stockage de données utilisant un système de refroidissement adiabatique bénéficient du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, Dans l'absolu, le refroidissement adiabatique semble être éligible au bénéfice du taux réduit, au regard des conditions fixées par l'article 21 de la proposition de loi, notamment compte tenu de ses bonnes performances énergétiques. Cependant, ce bénéfice ne serait pas automatique dans la mesure où d'autres conditions, qui n'ont pas trait au matériel lui-même, mais à la manière dont il est utilisé au sein du, sont exigées.

amendement tend à préciser expressément que les utilisant un système de refroidissement adiabatique bénéficieront du taux réduit, indépendamment des conditions exigées par l'article 21.

en rationalisant la consommation de foncier afin d'éviter la spéculation sur des terrains d'assiette potentiels, ainsi que la construction d'infrastructures laissées ensuite vacantes faute d'utilisateurs identifiés préalablement au lancement des projets. Ces pratiques gèlent des tènements qui pourraient être mis à profit par des acteurs engagés dans des démarches de fourniture effective de service. Lorsqu'elles conduisent à l'érection de pylônes dénués de tout équipement actif, elles aggravent l'impact environnemental lié à leur construction, qu'il s'agisse de la production de gaz à effet de serre, de l'artificialisation des sols, de l'impact visuel ou de la dégradation des paysages. Elles diminuent l'acceptabilité sociale de ce type d'équipements. La primauté de la protection de l'environnement sur la liberté d'établissement des acteurs économiques, actée par la Charte de l'environnement de 2004, qui en a fait un objectif de valeur constitutionnelle, trouve une application supplémentaire grâce à un déploiement d'infrastructures maîtrisé.

est ainsi libellé : La parole est à M. Éric Gold. Les administrations publiques doivent montrer l'exemple en matière de réduction de l'impact environnemental du numérique. Le premier levier consiste en une gestion responsable de l'équipement numérique. Le recours à une base de données, à la standardisation des terminaux, à la virtualisation et au permet non seulement de faire des économies de fonctionnement et de renforcer la sécurité informatique, mais aussi de gérer durablement les ressources numériques. Tel est l'objet de cet amendement qui vise à ce que les services de l'État, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements adoptent, une gestion optimisée, financière, fonctionnelle et durable de leur parc informatique et de l'ensemble de leurs moyens de communication. tend également à ce que les collectivités territoriales concernées par l'obligation d'établir une stratégie numérique durable évaluent l'impact environnemental des biens et services numériques qu'elles utilisent, en cohérence avec les dispositions prévues dans la proposition de loi pour les grandes entreprises.

dans les territoires. Celle-ci prévoit notamment de compléter le rapport au développement durable de ces collectivités par une stratégie numérique durable. La commission a donc émis un avis défavorable.

des politiques de couverture numérique du territoire et d'inclusion numérique. La répartition des sur le territoire constitue certes un enjeu important sur le plan environnemental, notamment en termes de consommation d'espace et d'énergie. ne nous semble pas relever de cet outil. La commission a fait le choix de privilégier les plans climat-air-énergie territoriaux comme outil de prise en compte de cette nécessaire planification territoriale des enjeux relatifs à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. La commission a donc émis un avis défavorable

The Shift Project indiquent que l'intensité énergétique de l'industrie numérique augmente au niveau mondial de 4 % par an. L'objectif de cette proposition de loi est de garantir la convergence entre la transition écologique et la transformation numérique et de veiller à ce que la transition numérique soit un accélérateur de la transition écologique. Nous sommes encore peu outillés pour faire de l'environnement un facteur déterminant dans nos choix politiques et stratégiques. La France manque d'outils et d'indicateurs partagés pour mesurer les impacts environnementaux du numérique et ainsi mieux cibler les actions à mettre en oeuvre prioritairement. Nous avons besoin de progresser collectivement sur l'évaluation environnementale de ce que nous mettons ou mettrons en place. Il apparaît donc nécessaire, avant de déployer des solutions numériques touchant essentiellement les secteurs de la mobilité, des télécoms, des voiries, notamment celles dites « smart

Comme nous l'avions souligné dans notre rapport, une solution numérique innovante n'est pas forcément vertueuse sur le plan de son empreinte environnementale. Les représentants de The Shift Project avaient d'ailleurs insisté sur ce point lors de leur audition. Cependant, plutôt qu'une réalisation systématique d'évaluation environnementale